et décembre 2020, trois ans se sont écoulés. Pendant ces trois années, le devis établi par l'État pour réaliser cette déviation est passé de 48 millions d'euros à 81 millions d'euros, soit une augmentation de 65 %.

l'hypothèse d'une deuxième phase qui commencerait en 2023. En effet, 2023 devait être la date d'achèvement de la déviation selon l'accord de cofinancement de janvier 2018

sont inscrits à ce titre dans l'actuel contrat de plan État-région pour un montant de 48 millions d'euros, dont 27,5 millions d'euros sont pris en charge par l'État. Cet engagement a été confirmé dans le cadre du projet de développement de territoire qui accompagne le projet Cigéo. Depuis, plusieurs étapes ont été engagées. Les acquisitions foncières nécessaires aux travaux ont été réalisées en quasi-totalité. La dérogation espèces protégées, après avis du Conseil national de la protection de la nature, et l'autorisation au titre de la loi sur l'eau ont été obtenues ; elles ont fait fait l'objet des prolongations nécessaires à la fin de l'année 2020. Les premiers travaux vont donc pouvoir débuter, avec le lancement de la première phase intégrant, notamment, les travaux du giratoire de Tronville. Par ailleurs, 4 millions d'euros supplémentaires seront affectés cette année pour réaliser les fouilles archéologiques préventives. Vous l'avez mentionné, l'actualisation des études détaillées par le maître d'oeuvre chargé de la finalisation du dossier a fait apparaître une augmentation importante du coût de l'opération, à hauteur de 33,5

et de reprise de calcul des fondations. Les fouilles archéologiques très importantes rendues nécessaires par la découverte d'une nécropole ont fortement contribué au renchérissement du coût de ce projet.

complémentaire nécessaire à cette seconde phase devra donc être recherchée dans le cadre de la prochaine contractualisation sur les infrastructures, qui prendra effet à compter de 2023. Je vous confirme que l'État reste particulièrement mobilisé sur ce dossier.

Cette société souhaite exploiter du gaz de couche jusqu'en 2040, ce qui pose à mon sens deux problèmes majeurs : cela ne concourt pas à la réussite de notre stratégie bas-carbone et c'est l'illustration d'un droit minier déconnecté du droit environnemental. Cette concession couvrirait près de 200 kilomètres carrés et toucherait quarante communes. quarante et une plateformes de forage. Pour un projet aussi impactant, une simple enquête publique a eu lieu en septembre 2020, à laquelle seules quatorze communes ont eu les moyens de répondre. Des associations et beaucoup d'élus locaux s'opposent à ce projet, qui aurait un impact économique limité et constituerait une menace pour la biodiversité, les sols et la ressource en eau. Surtout, la société n'a pas convaincu qu'elle avait les capacités techniques et financières suffisantes pour exploiter ces hydrocarbures sans recours à la fracturation hydraulique, interdite depuis 2017. La demande de concession relevant du droit minier, elle échappe totalement au code de l'environnement. Elle n'a donc pas fait l'objet d'une concertation préalable ou d'un débat public, et aucune évaluation environnementale n'a été exigée. Ces anomalies sont difficilement compréhensibles. L'étude d'impact du projet de loi Climat et résilience a souligné que le droit minier prend mal en compte les enjeux économiques, environnementaux et sociaux et la participation du public. Une commission d'enquête du Sénat a recommandé, dans son rapport de septembre 2020, de mettre un terme aux asymétries entre le code minier et le code de l'environnement. Pourtant, la société La Française de l'énergie va sans doute profiter du droit de suite. Ma question est donc la à l'heure où un début de réforme du code minier apparaît dans le projet de loi Climat et résilience, est-il raisonnable d'autoriser une concession de gaz de couche sans évaluation environnementale ni véritable débat citoyen ? Est-il cohérent d'autoriser pour vingt ans encore l'extraction de ressources fossiles d'hydrocarbures à à rebours de nos engagements climatiques

Cette demande est actuellement en phase d'instruction locale et a été soumise à enquête publique du 10 septembre au 13 octobre 2020. L'instruction de la demande se poursuivra par une phase d'instruction nationale qui, en application des des dispositions du code minier, concernera l'appréciation des capacités techniques et financières du demandeur pour mener à bien les travaux d'exploitation et assumer les obligations pour préserver les intérêts de sécurité du travail, de sécurité des édifices publics ou privés

Comme vous l'indiquez, la loi du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures a posé le principe du maintien des titres en cours de validité et la possibilité d'octroi de concessions, exclusivement dans le cadre du droit de suite d'un permis exclusif de recherches.

si la concession est octroyée au pétitionnaire, les enjeux environnementaux seront pris en compte avec la plus grande attention lors de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux miniers nécessaires pour réaliser l'exploitation. l'exploitation. Comme vous l'avez rappelé, la réforme du code minier prévue par le projet de loi Climat et résilience ira plus loin, en introduisant notamment l'obligation de réaliser une analyse environnementale, économique et sociale pour l'octroi et l'extension des titres miniers d'exploration et d'exploitation. Les mêmes modalités s'appliqueront à la prolongation des titres exclusifs d'exploitation et des transformations de titres exclusifs de recherches en titres exclusifs d'exploitation. Dans le cadre du débat démocratique que nous souhaitons voir renforcé, le demandeur d'un titre minier mettra à disposition du public sur un site internet son dossier de demande, ainsi que la réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable et à l'avis économique et social du Conseil général de l'économie avant l'ouverture de l'enquête publique ou la réalisation de la participation du public, toutes deux prévues au code de l'environnement. Enfin, les collectivités territoriales, communes et éventuellement établissements publics intercommunaux, seront systématiquement consultées tout le long de la vie du titre minier, du dépôt de la demande à la fermeture des installations.

doit pouvoir être saisie d'un projet de cette envergure. Il n'est plus compréhensible, après les accords de Paris, que la région Lorraine et l'avenir de notre climat soient encore impactés par un projet aussi toxique.

En effet, ce décret impose de nouvelles normes aux EPCI chargés de l'aménagement et de la gestion de ces aires, y compris à ceux qui ont déjà rempli leurs obligations en créant une aire de grand passage sur leur territoire. Ainsi, la mise en place d'une norme de superficie de 4 hectares- excusez du peu ! -est particulièrement problématique dans le contexte de tension foncière de certains départements, dont celui du Bas-Rhin, qui est le mien. qui est le mien. Cette superficie, d'ailleurs désapprouvée en son temps par les représentants locaux des gens du voyage siégeant à la commission départementale consultative, est de nature à favoriser la constitution de groupes dont la taille entraînera inévitablement des difficultés de gestion et de cohabitation.

Vous le savez, les aires de grand passage ne bénéficient d'aucune aide en fonctionnement et les seules aides à l'investissement n'interviennent qu'à travers la DETR. En conséquence, quelles aides l'État peut-il apporter aux EPCI pour résoudre ces difficultés ? Est-il envisageable d'apporter une modification au décret concerné ?

vous avez souhaité appeler l'attention de la ministre du logement sur la portée des normes issues du décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 relatif aux aires de grand passage. Ce décret répond à l'objectif général visé par le législateur depuis 2000 de permettre l'accueil temporaire des gens du voyage. Il s'appuie aussi sur des constats partagés lors de plusieurs concertations avec des collectivités territoriales, leurs associations et des représentants des usagers, ainsi que des travaux techniques de la Commission nationale consultative des gens du voyage. Ce décret fixe des conditions minimales d'accueil, formule des recommandations et laisse aux communes et aux EPCI le soin d'adapter ces dispositions aux réalités locales, par exemple concernant le règlement du droit d'usage et de la tarification des prestations qui peut faire l'objet d'un forfait. Il prévoit également des dérogations pour tenir compte des disponibilités foncières, des spécificités topographiques ou des besoins particuliers définis par le schéma départemental. L'expérience montre que, lorsque les aires de grand passage prévues par le schéma départemental ont été réalisées, la majorité des installations se déroulent dans des conditions sereines et les stationnements illicites sont moindres. C'est précisément l'un des objectifs prioritaires du schéma départemental du Bas-Rhin 2019-2024. Sur les quatre aires de grand passage initialement prévues, deux seulement sont en service. Le schéma prescrit donc la réalisation de ces deux aires afin d'améliorer l'accueil. Il prévoit également un diagnostic spécifique sur les grands passages dans le cadre d'une concertation avec les EPCI concernés et des propositions d'aménagement.

pour un coût prévisionnel de l'opération porté à 475 392 euros, soit un taux d'aide de près de 60 %. Cet équipement, qui avait été prescrit par le précédent schéma, est par ailleurs cofinancé par la communauté de communes du Pays de Niederbronn-les-Bains. D'autres financements peuvent être accordés tels que la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL, ou le Fonds européen de développement régional, le Feder. Un cofinancement de plusieurs collectivités peut également être envisagé pour un équipement en gestion mutualisée.

Elle fait partie des départements dont les sols dits « argileux » déstabilisent et fissurent les constructions. Les propriétaires de maisons et bâtiments endommagés se trouvent dans une situation catastrophique, dans l'impossibilité financière de réaliser les réparations des dommages provoqués par les mouvements des sols, de louer un autre logement et encore moins de vendre leur bien déprécié. Quant aux maires des communes concernées, ils ont été et sont encore dans une grande solitude pour accompagner les propriétaires. Certaines communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle, pas toutes, tant s'en faut, sans qu'élus et population comprennent toujours pourquoi. Les services de l'État n'ont pas de réponse précise et concrète à leur apporter. En 2019, une mission d'information du Sénat a travaillé sur le sujet de la gestion des risques climatiques et de l'évolution des régimes d'indemnisation. Une proposition de loi a été déposée et adoptée à l'unanimité le 15 janvier 2020, mais elle n'a pas été inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ! Depuis, la loi de finances pour 2021 a prévu un dispositif d'aide exceptionnel, actuellement mis en oeuvre les préfectures. les conditions posées à l'indemnisation sont très restrictives, imposant des limitations de délai d'achèvement de la construction et de date de dépôt de demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Enfin, l'indemnisation ne vise que les propriétaires très modestes au sens des plafonds de ressources de l'ANAH. de l'ANAH. Le Gouvernement entend-il ces propriétaires victimes des catastrophes naturelles de ces dernières années et que leur répond-il ? L'aide exceptionnelle ne va toucher qu'un nombre réduit de propriétaires : vers qui la très grande majorité d'entre eux devra-t-elle se tourner ? Quels outils le Gouvernement prévoit-il pour que les maires se sentent épaulés ? Ils s'inquiètent en effet du coût des études de sols qu'ils ont demandées. Ils craignent également que leur responsabilité ne soit engagée en cas d'effondrement des maisons. Que leur répond le Gouvernement ?

de ce fonds d'urgence, le Gouvernement, en application de la loi ÉLAN et par arrêté du 22 juillet 2020, a pris des mesures préventives concernant les constructions neuves, en imposant des études géotechniques dans les zones d'aléas pour le retrait-gonflement d'argile. Il s'agit de s'assurer que ce type de dégâts ne se reproduise pas pour les constructions à venir. Pour remédier à certaines situations d'urgence liées à la sécheresse de 2018, la loi de finances pour 2020 a prévu la mise en place exceptionnelle, à hauteur de 10 millions d'euros, d'un dispositif de soutien aux victimes les plus affectées par l'épisode. Le phénomène de retrait-gonflement des sols survenu en 2018 implique un total de 5 680 communes, qui ont demandé une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ; 3 981 d'entre elles ont reçu un avis favorable et ne sont donc pas concernées par ce dispositif exceptionnel d'urgence. Les 1 699 demandes avec un avis défavorable de la commission correspondent à environ 15 000 bâtiments. Les dommages visés impliquent des travaux lourds et coûteux, portant sur la structure ou les fondations. D'une manière générale, il apparaît que, dans le cas des dossiers pris en charge par le dispositif de catastrophe naturelle, le montant des travaux réalisés à la suite d'un sinistre lié au phénomène de retrait-gonflement des argiles est supérieur à 25 000 euros. Il est donc nécessaire, dans le cas de ce dispositif exceptionnel, de cibler prioritairement les propriétaires aux revenus modestes, qui se trouveraient, sans cette aide, dans l'impossibilité de réaliser de tels travaux. La typologie des demandes reçues depuis la mise en place de ce fonds conduit à étudier son ouverture à des ménages aux revenus intermédiaires. Ce point fait l'objet d'un travail interministériel. Plus largement et à plus moyen terme, il apparaît que le régime de catastrophe naturelle est un dispositif ancien dont les critères peinent à s'adapter parfaitement au contexte de multiplication des sécheresses et de leurs conséquences sur le bâti existant. Le Gouvernement est déterminé à traiter les conséquences de ces phénomènes et a missionné l'IGF, l'IGA et le CGEDD pour faire un diagnostic et des propositions. Les conclusions de la mission sont attendues au printemps. Certaines de ces propositions pourraient être intégrées dans la proposition de loi Baudu, portant sur ce sujet, qui doit désormais être examinée au Sénat. La parole est à M. Jean Pierre Vogel, pour la réplique. Je vous remercie de cette madame la secrétaire d'État, mais j'espérais avoir des informations plus satisfaisantes. Le Gouvernement a commandé de nouvelles études, alors que tout est dans le rapport sénatorial Bonnefoy-Vaspart de 2019. C'est sans doute la volonté politique qui manque, sans doute aussi peut-être les moyens financiers ... Le Gouvernement ne peut ignorer plus longtemps le sujet et rester sourd aux doléances et à la souffrance de ces propriétaires.

Longtemps considérée comme abondante, elle est aujourd'hui perçue comme un bien limité à la qualité menacée. Parmi les nombreux défis de développement durable, l'accès à l'eau est donc fondamental. La loi NOTRe a modifié les règles de la compétence « eau et assainissement ». Ainsi, les établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, devront d'ici au 1 janvier 2026 prendre le relais des communes. À cette date, les communes déjà raccordées et celles qui ne le sont pas

Le rendement est évalué à 80 %, c'est-à-dire qu'entre l'eau pompée et celle qui est distribuée, 20 % de l'eau est perdue dans le transport, à savoir 17 millions de mètres cubes. Les remises à niveau nécessaires des réseaux d'eau et d'assainissement au sein des EPCI nécessitent des investissements colossaux. Si les communes ont pu bénéficier des aides de l'Agence de l'eau, du département, de la région, avec des taux de subvention atteignant 80 %, la situation a bien changé, et ces taux sont aujourd'hui divisés par deux. Certaines communes ont été des modèles en devançant les intercommunalités. Elles ont emprunté pour construire leur réseau d'assainissement communal. Ainsi, dans une intercommunalité, certaines villes ont un réseau d'assainissement, d'autres non. L'idée est donc de trouver un équilibre entre bonne gestion et solidarité, afin de ne pas pénaliser les bons élèves au sein d'une même intercommunalité. Le renouvellement des conduites d'eau potable et des réseaux d'assainissement ayant un impact très important sur l'économie de la ressource et la préservation des milieux naturels, l'Association des maires ruraux de Seine-et-Marne a émis l'idée qu'une partie des crédits verts européens soit dédiée à la rénovation des réseaux, permettant ainsi d'éviter une forte augmentation des prix à la charge du contribuable.

prise en compte de nouveaux enjeux comme l'adaptation au changement climatique et la lutte contre l'érosion de la biodiversité. Les instances de gouvernance des agences de l'eau regroupant l'ensemble des acteurs ont été amenées à faire des choix et, par conséquent, à mettre davantage de sélectivité dans les conditions d'octroi des aides. Les interventions des agences de l'eau ont été recentrées, d'octroi des aides. Les interventions des agences de l'eau ont été recentrées, dans une logique de solidarité territoriale, sur les collectivités qui rencontrent de façon structurelle des difficultés pour faire face aux investissements relatifs aux équipements d'infrastructures. Ainsi, pour la période 2019-2024, 2019-2024, ce sont 4,5 milliards d'euros d'aides qui seront engagés par les six agences de l'eau en faveur de projets d'installation de traitement, de renouvellement de réseaux ou d'interconnexion. La gestion des eaux pluviales bénéficie d'une enveloppe dédiée de 850 millions d'euros. À titre d'exemple, l'agence de l'eau Seine-Normandie a d'ores et déjà engagé 238 millions d'euros en 2019 et 226 millions d'euros en 2020 en faveur d'infrastructures dédiées au petit cycle de l'eau. En complément de ces crédits, les agences de l'eau vont engager dans le cadre du plan de relance, dès 2021, 250 millions d'euros d'aides pour des projets portant sur la modernisation du réseau d'eau potable, sur la mise aux normes de stations de traitement des eaux usées, sur la rénovation des réseaux d'assainissement, y compris les mauvais branchements, sur le déraccordement des rejets d'eaux pluviales et leur infiltration à la source, ainsi que sur l'hygiénisation des boues d'épuration. L'actualité récente nous montre combien ces travaux sont d'importance. Sur ce montant global de 250 millions d'euros de crédits du plan de relance en faveur de ces mesures, une enveloppe de 68 millions d'euros est allouée à l'agence de l'eau Seine-Normandie. Les projets qui pourront bénéficier de ces crédits sont pour la plupart identifiés et leur répartition est équilibrée par région et par département.

dans une interview du 31 janvier dernier, le ministre des transports, Jean-Baptiste Djebbari, a déclaré : « Quand les moyens sont là avec une bonne qualité de service et la bonne offre commerciale, il y a une clientèle pour les trains de nuit. » Fort de cette réalité, des enjeux écologiques et des opportunités de financement ouvertes par les plans de relance français et européen, le Gouvernement a fait le choix de développer de nouvelles lignes de trains de nuit. Je soutiens bien évidemment cette orientation, mais je veux vous alerter sur la nécessité absolue de tenir compte, dans vos choix, des besoins en matière d'aménagement du territoire et de l'insuffisance de transports dans certains départements.

de développement des trains de nuit, notre région ne bénéficie pas d'une remise en service du train de nuit Aurillac-Paris, alors même qu'Aurillac est la préfecture de France métropolitaine la plus éloignée d'un axe autoroutier. Or les éléments diffusés en amont de la publication du rapport du Gouvernement sur ce sujet ne nous rassurent pas vraiment. Aussi, pouvez-vous m'assurer,

En tant qu'ancienne rapporteure de la loi d'orientation des mobilités, j'y étais- vous le savez -très attachée. Nous poursuivons, et amplifions même, cette dynamique dans le plan de relance, puisque la priorité a été réorientée vers le développement du ferroviaire, là où des gouvernements précédents- vous le savez également

Paris-Nice pour le printemps 2021 et de la ligne Paris-Tarbes pour 2022, avec un prolongement vers Lourdes, Dax et Hendaye en haute saison. Les modalités de reprise sont en train d'être précisées par la SNCF. Nous savons combien les attentes des voyageurs et des élus Enfin, il nous faut penser le maillage de demain. Le ministre Djebbari a indiqué que près de dix lignes de trains de nuit pourraient voir le jour d'ici à 2030. Un rapport devrait être prochainement remis au Parlement, conformément aux engagements de la loi d'orientation des mobilités votre serviteur- et je m'en félicite. Dans le cadre de la réalisation de ce rapport, nous avons pris note des fortes demandes des élus du Cantal en faveur d'un train de nuit desservant Aurillac. Je sais que ce sujet vous est particulièrement important. Le rapport qui sera remis s'attache à définir des corridors. Il s'agira ensuite de poursuivre les échanges avec les opérateurs pour affiner les tracés qui soient les plus pertinents, afin d'acheter les matériels roulants nécessaires. Monsieur le sénateur, je peux d'ores et déjà vous indiquer qu'Aurillac fait bien partie des hypothèses de desserte examinées dans cette étude, depuis le corridor reliant Paris à Toulouse. Nous aurons donc l'occasion de poursuivre ces échanges lors des débats à venir au Parlement, et le Gouvernement répondra toujours présent s'agissant de cet enjeu majeur de désenclavement de nos territoires et de décarbonation de nos modes de transport.

de rétablir de l'équité territoriale dans les politiques publiques et d'adresser des messages d'espoir à la ruralité. Le déploiement des trains de nuit en est l'occasion. Nous comptons sur vous, et vous imaginez bien que nous suivrons ce dossier avec la plus grande détermination. Je vous remercie encore une fois de votre réponse, qui nous ouvre donc des perspectives positives. La parole

explique que certains ouvrages nécessitent des réparations lourdes ou soient démolis alors même qu'ils n'ont que quarante ou cinquante ans d'existence. Dès lors, il est nécessaire d'entreprendre des actions, comme le maintien en bon état des étanchéités pour éviter des infiltrations d'eau, des joints de chaussée, la peinture des parties métalliques pour éviter leur corrosion ou la dévégétalisation. Ces actions sont essentielles pour maintenir, voire prolonger, la durée de vie des infrastructures. Nous constatons, hélas, un manque d'investissement de l'État, mais aussi des collectivités territoriales. Nous devons également déplorer un manque de compétences techniques avec, notamment, la difficulté pour les départements de recruter des ingénieurs spécialisés dans les ouvrages d'art. Si l'État est doté d'un référentiel technique pour la gestion des ponts, qui prévoit un cycle de visites régulières, la méthode d'évaluation des ponts repose sur une inspection visuelle, qui ne permet de suivre que les dégradations visibles. Elle est donc insuffisante. Nous constatons tous que nos communes se retrouvent à devoir supporter des charges incombant à l'entretien de ces ouvrages d'art sans pour autant bénéficier des moyens techniques et financiers nécessaires. C'est le cas dans onze communes membres de la communauté de communes de de Flandre intérieure traversées par la ligne à grande vitesse Nord. La jurisprudence constante en la matière pose le principe selon lequel « la domanialité et la propriété d'un pont sont celles de la voie portée par l'ouvrage Aujourd'hui, SNCF Réseau exige l'application stricte de cette jurisprudence. C'est d'autant plus dommageable que les joints de chaussée sont des dispositifs complexes, dont la qualité de conception et de mise en oeuvre conditionne directement le bon fonctionnement et la pérennité des ouvrages d'art et non de la voie circulante. Les communes doivent donc prendre en charge des ouvrages de rétablissement des voies dont elles sont propriétaires, alors même que ces ouvrages ont été construits pour permettre de nouvelles infrastructures. Or cette prise en charge excède bien souvent leurs capacités financières. Le législateur a pris conscience de ce problème. En effet, la loi du 7 juillet 2014 vise à repartir les responsabilités et les charges financières concernant les ouvrages d'art de rétablissement des voies. De même, un arrêté du 22 juillet 2020 a pour objet de recenser les ouvrages ayant rétabli des voies de communication des collectivités territoriales interrompues par une voie de l'État ou de ses opérateurs. Or les ouvrages de rétablissement surplombant une voie du réseau autoroutier concédé sont exclus du recensement, car la source de l'obligation pour les sociétés concessionnaires de négocier avec les collectivités territoriales des conventions de gestion se trouve dans la convention de concession elle-même. Aujourd'hui s'ouvre une phase de négociation de conventions par lesquelles l'État et ses établissements publics perdront en charge, dans les conditions prévues par la loi, une partie des frais liés à la surveillance et l'entretien de ces ouvrages. La conclusion de ces conventions est une opportunité pour les onze communes de la communauté de communes de Flandre intérieure, car celles-ci définiront la répartition de frais d'entretien des ouvrages avec, notamment, une prise en compte des capacités financières.

par les services de l'État et de ses opérateurs de recensement des ouvrages d'art de rétablissement ne faisant pas l'objet de conventions, dont les ponts-routes. Il s'agissait d'un travail inédit, qui a abouti, après une concertation organisée avec les collectivités territoriales sur la base d'un recensement provisoire, à la publication d'une liste de 9 480 ouvrages d'art, dont plus de 4 4 000 sont situés au-dessus du réseau ferré français. En complément de cette liste, le ministère des transports va très prochainement mettre en place un formulaire de contact, afin que les collectivités puissent soumettre des ouvrages d'art de rétablissement dont elle n'avait pas pu soumettre la situation lors du recensement initial. Ces ouvrages d'art feront progressivement l'objet de conventions sur une période qui, en raison du nombre d'ouvrages à conventionner, conventionner, s'étalera sur un temps long. Une priorisation du conventionnement des ouvrages sera nécessaire. Au vu de la disparité des réseaux concernés, en termes de nombre d'ouvrages et de caractéristiques techniques, il apparaît préférable que l'État et ses opérateurs définissent chacun la politique de priorisation de conventionnement des ouvrages situés au-dessus de leur réseau, l'État veillant à la cohérence de l'ensemble. Ainsi, SNCF Réseau travaille actuellement avec les collectivités territoriales ayant sollicité le gestionnaire pour définir le périmètre et le contenu des conventions de gestion. Ces conventions s'inscriront dans le cadre défini par le code général de la propriété des personnes publiques, lequel dispose que le « principe de référence », donc la prise en charge par le gestionnaire de la « nouvelle » infrastructure de l'ensemble des charges relatives à la structure de l'ouvrage, bénéficie, sauf accord contraire des parties, aux collectivités locales propriétaires d'un ouvrage de rétablissement dont le potentiel fiscal est inférieur à 10 millions d'euros. Vous pouvez compter, monsieur le sénateur, sur notre pleine mobilisation pour la mise en oeuvre

ils nous disent combien leurs relations avec la SNCF sont à tout le moins défaillantes, lorsqu'elles ne sont pas inexistantes. Je ne parle pas de la gestion des gares ; je vous

tout d'abord à m'associer et associer le Gouvernement aux pensées émues adressées à la famille et aux proches d'Olivier Dassault, notre collègue de l'Assemblée nationale disparu dans les circonstances dramatiques que nous savons. Vous m'interrogez sur les actions de communication qui peuvent être menées par la SNCF, notamment à l'intention des maires, en cas d'incident. La loi pour un nouveau pacte ferroviaire a transféré depuis le 1 janvier 2020 à SNCF Réseau la coordination en matière de gestion de crise. Il est Il est ainsi prévu que « SNCF Réseau a pour mission d'assurer [ ...] des missions transversales nécessaires au bon fonctionnement du système de transport ferroviaire national, au bénéfice de l'ensemble des acteurs [ ...], notamment en matière de gestion de crise et de coordination des acteurs pour la mise en accessibilité du système de transport ferroviaire national aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ». Il revient donc à la SNCF, en cas d'incident, de coordonner les différents acteurs du système ferroviaire en vue de rétablir la situation d'exploitation normale. Dans ce contexte, le plan d'intervention et de sécurité, qui doit être activé en cas d'événement important, est établi par le gestionnaire d'infrastructure chargé de la gestion opérationnelle des circulations, en concertation avec les autorités administratives compétentes et, le cas échéant, les autres gestionnaires d'infrastructures chargés de l'exploitation aux interfaces, conformément à l'article 46 du décret n° 2019-525 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires. Par ailleurs, il est envisagé d'équiper de nombreux passages à niveau d'une pancarte portant l'inscription d'un numéro d'appel pour permettre aux usagers de joindre les services opérationnels de SNCF Réseau en cas de dysfonctionnement. le ministre Djebbari indique par ailleurs qu'il rappellera à la SNCF, après votre sollicitation, l'importance de ces dispositions. Nous partageons avec vous la nécessité de bien associer les élus locaux, notamment dans le cadre de la gestion des incidents et, plus globalement, de l'évolution de l'offre ferroviaire.

la ligne des chemins de fer de Provence, ou train des pignes pour les plus nostalgiques. Une ligne qui, avec ses salariés, a connu des coups durs, notamment à la suite des récentes intempéries, et qui s'est toujours relevée. La région Sud est concessionnaire, depuis le 1 janvier 2007, de cette ligne qui est exploitée par une régie, dans le cadre d'un contrat de délégation de service public de dix ans. Cette ligne aux 58 circulations par jour bénéficie d'investissements importants réalisés par la région Sud et l'État depuis des années en matière d'infrastructures et de gares ; elle sera bientôt dotée de matériels neufs pour près de 56 millions d'euros. Cette ligne demeure une ligne de vie structurante d'aménagement du territoire et un vecteur touristique fort pour nos vallées du moyen et haut pays. Les communes traversées ou limitrophes de cette ligne atypique attendent le transfert de pleine propriété de l'État à la région pour l'euro symbolique, un transfert qui permettrait le développement du transport ferré dans ces territoires, mais également, et surtout, des projets de valorisation économique du patrimoine.

La région Sud a en effet adressé en 2018 une demande de transfert de propriété à laquelle le ministère des transports a répondu favorablement. Le transfert reste toutefois subordonné à la signature d'une convention entre l'État et la région, qui est en cours de rédaction. Cette convention doit préciser la date à laquelle le transfert intervient, la nature des biens transférés et les conditions financières et techniques du transfert. Les services de l'État et de la région ont arrêté un projet de convention. Après la réunion qui s'est tenue le 8 février 2021 entre les services de l'État et ceux de la région, des précisions doivent encore être apportées sur le périmètre des parcelles concernées et sur la valorisation des actifs transférés préalablement à la signature de la convention par le président de région et le préfet. Ces précisions techniques apportées, le transfert pourra être concrétisé en bon ordre, puisqu'il y a un accord de principe de l'État et de la région sur ce point. monsieur le sénateur, l'État et les collectivités travaillent main dans la main pour redynamiser les lignes de desserte fine du territoire, qui contribuent à des transports plus propres pour les déplacements du quotidien de nos concitoyens et assurent un maillage territorial essentiel. Ce sont 6,5 milliards d'euros qui devraient être investis

quelques semaines après son élection à la présidence de la République, Emmanuel Macron inaugurait la voie nouvelle entre Rennes et Connerré, permettant de mettre Rennes à une heure

compte tenu de la difficulté actuelle à mobiliser des fonds, soit des opérations plus ponctuelles permettant d'améliorer, à la fois, la sécurité routière et l'accessibilité de la Bretagne occidentale.

le plan de relance pourrait opportunément servir de moyen de financement. Je souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière et les perspectives d'investissement que l'on peut attendre pour ces deux lignes, entre Rennes et Brest, d'une part, et entre Rennes et Quimper, d'autre part.

de 2018, à améliorer l'accessibilité ferroviaire de la pointe finistérienne. Cet objectif a été confirmé dans la loi d'orientation des mobilités de 2019. prévoit le lancement d'études pour une ligne nouvelle entre Rennes et Redon, créant une liaison performante, proche d'une heure, entre Rennes et Nantes. Ce projet doit permettre, à la fois, d'améliorer les transports du quotidien et de rapprocher le temps de trajet entre Quimper et Paris de l'objectif des trois heures. Ainsi, le ministre a demandé en février 2020 d'élaborer une feuille de route pour le grand projet de liaisons nouvelles Ouest Bretagne-Pays de la Loire. Celle-ci sera rédigée sur la base d'une actualisation des études réalisées pour le débat public en 2014 et 2015, ainsi que pour l'étape complémentaire qui lui a succédé en 2016 et 2017. Il s'agit désormais d'agir sur les deux axes bretons. Pour l'axe Nantes-Rennes-Finistère sud, l'objectif est de lancer les études préliminaires pour la réalisation d'une ligne nouvelle entre Rennes et Redon et permettre la desserte à la demi-heure entre Nantes et Rennes avec l'amélioration de la ligne existante entre Nantes, Savenay et Redon. Pour l'axe nord Rennes-Brest, un schéma directeur d'axe visant une amélioration amélioration progressive des infrastructures est en cours, avec l'objectif de mettre à terme Brest à trois heures de Paris. Ce schéma directeur décrira les solutions d'infrastructures et de services à mettre en oeuvre à différents horizons, au regard des besoins de mobilité. Parmi les aménagements envisagés, des relèvements de vitesse à plus de 160 kilomètres par heure sur certaines sections de la ligne classique nécessiteront à terme la suppression des passages à niveau sur celles-ci. S'agissant enfin du passage à niveau du Relecq-Kerhuon, celui-ci a été retiré en 2001 du plan de sécurisation national des passages à niveau, condition pour que l'État envisage de participer financièrement à sa suppression. L'instance nationale des passages à niveau peut à tout moment examiner l'opportunité d'y inscrire de nouveau ce passage s'il apparaît qu'il remplit les conditions de trafic et d'accidentologie. La parole

le 15 décembre 2020, à l'Assemblée nationale, le Premier ministre a déclaré que le Gouvernement n'avait pas l'intention d'affaiblir ou de démanteler EDF. Pourtant, les activités d'EDF seront dorénavant réparties entre plusieurs entités de statuts différents. EDF Azur serait l'entreprise qui s'occuperait des barrages hydroélectriques. Le Sénat a déjà déploré le manque de transparence du Gouvernement sur ce projet structurant pour l'avenir de la souveraineté et de la transition écologiques du pays. Or le démantèlement s'inscrit dans un contexte particulier avec la mise en concurrence des concessions hydrauliques, sous la pression de la réglementation européenne. Cependant, les concessions hydrauliques et l'économie hydroélectrique contribuent depuis des décennies à l'aménagement des territoires ruraux. Cet enjeu est donc crucial pour les collectivités territoriales et leurs territoires. Par exemple, EDF hydraulique Lot-Truyère représente 20 barrages, qui alimentent 15 centrales. Les aménagements des vallées du Lot et de la Truyère produisent ainsi 10 % de l'énergie hydroélectrique en France. Ces centrales sont donc d'un intérêt national. Or Mme Pompili avait déclaré que la préservation de l'intérêt national pourrait se faire dans le cadre d'une prolongation ou d'une nouvelle concession. Ma question porte donc sur la stratégie du Gouvernement, qui s'abrite, trop souvent, derrière les contraintes européennes pesant sur le projet pour ne pas dévoiler sa position. Pour être plus précis, Mme Pompili avait déclaré, il y a deux ans, au Sénat, que « le traitement des concessions hydroélectriques dans la vallée du Lot et de la Truyère s'inscrira dans la réponse globale et équilibrée recherchée avec la Commission européenne. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Malheureusement, cette réponse convenue laisse dans l'expectative la population de la vallée du Lot et de la Truyère. Aussi, pouvez-vous, madame la secrétaire d'État, préciser les intentions du Gouvernement s'agissant de la prorogation des concessions du Lot et de la Truyère ? Allez-vous prolonger ces concessions ? Quelles conséquences la création d'EDF Azur aura-t-elle sur les milliers d'emplois concernés ? Il est essentiel que le Gouvernement s'engage fermement pour que sa politique économique ne connaisse pas une nouvelle déconvenue, semblable à celle qui fait suite à l'annonce de la suppression de 750 emplois dans l'usine Bosch d'Onet-le-Château,

activement à résoudre le contentieux engagé par la Commission européenne, portant notamment sur l'absence de renouvellement par mise en concurrence des concessions hydroélectriques échues. Cette situation nuit aux investissements dans le secteur et est source d'inquiétude- je vous rejoins sur ce point -pour les entreprises, les salariés et les collectivités. Dans le même temps, vous le savez, une réflexion sur la réorganisation sur la réorganisation du groupe EDF, projet dit « Hercule », est en cours. Ce projet de réorganisation est plus vaste que la seule activité hydroélectrique d'EDF puisqu'il concerne toutes les activités du groupe. C'est dans ce contexte de contentieux européen et de réflexion sur l'organisation du groupe EDF que le Gouvernement explore plusieurs scénarios pour le renouvellement des concessions, dont celui de l'attribution à une structure publique. Mais, j'insiste, rien n'est arrêté et aucune décision n'a été prise. Les échanges avec la Commission européenne se poursuivent. Le Gouvernement recherche une réponse globale et équilibrée pour l'exploitation de l'hydroélectricité en France. La vision et les engagements du Gouvernement sont clairs : la solution retenue devra permettre la pérennisation et le développement du parc hydraulique français. L'hydroélectricité est en effet absolument cruciale pour notre transition énergétique, mais également pour la gestion de la ressource en eau. C'est donc une activité essentielle dans le contexte du changement climatique. Vous l'avez rappelé, elle contribue également significativement à l'économie locale. Nous serons, comme vous, attachés à la préservation des personnels des sociétés exploitantes. La parole

Si l'objectif consistant à développer de telles énergies est largement partagé, il n'en demeure pas moins que les modes de production de celles-ci ne sont pas sans impact pour les populations environnantes- nuisances esthétiques, sanitaires ou encore olfactives

Il est donc nécessaire que ces installations soient réalisées en accord avec les habitants et les élus des territoires concernés, au premier rang desquels figurent les maires. Ce n'est malheureusement pas le cas ; très souvent, ces projets sont menés sans l'accord des élus concernés. Les tensions vont s'accroître, puisque l'accélération du développement des énergies renouvelables est inscrite dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, avec, d'ici à 2028, le doublement de la production d'électricité éolienne et la création de 7 000 mâts supplémentaires. Cette

Des projets d'installation de méthaniseurs sont également source d'une inquiétude réelle dans nos territoires. Dans ce contexte, il semble donc indispensable de donner la capacité aux élus municipaux de s'opposer à de telles réalisations

2019, elle a permis d'éviter l'équivalent des émissions de près de 8 millions de véhicules, tout en couvrant plus de 7 % de la consommation électrique française. Ensuite, la filière a permis de créer plus de 20 000 emplois directs ou indirects en France. Vous souhaitez, et je vous rejoins en cela, que les élus participent, avec plus de pouvoir, à la planification du développement de l'éolien et de la méthanisation, en ayant un droit de regard sur ces projets. L'implication des collectivités territoriales dans le développement des énergies renouvelables est absolument indispensable renforcement de la résilience face à ses effets, qui est en cours d'examen, une déclinaison par région des objectifs d'énergies renouvelables de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE). Cette nouvelle disposition permettra, en concertation avec les régions et les collectivités, de répartir les objectifs de développement de chaque énergie renouvelable, y compris l'éolien et la méthanisation, en fonction des potentiels et des spécificités de chaque territoire et de chaque région. Avec la définition de tels objectifs régionalisés de développement de ces énergies, les territoires disposeront d'une plus grande visibilité, à leur échelle, pour ce qui concerne tant les besoins que les possibilités de développement de ces énergies. En outre, la réglementation garantit déjà l'implication des élus locaux lors du processus d'autorisation d'une installation éolienne ; leur avis est systématiquement demandé lors de l'enquête publique. La loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, dite ASAP,

pour associer encore plus les collectivités aux phases préliminaires de ces projets. Enfin, je souligne que les documents locaux d'urbanisme qui sont à la main des élus locaux, tels que les schémas de

-sur l'installation d'équipements qui posent un problème en matière de qualité de vie de leurs habitants et d'attractivité de leur commune ? Vous n'avez pas répondu à cette question. Vous m'avez rappelé la réglementation et l'intérêt des énergies renouvelables ; c'est très bien, mais là n'est pas la question.

Nous vous savons très attentif, monsieur le ministre, à la défense des intérêts de l'agriculture, dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune (PAC). Le cadre budgétaire obtenu est plutôt satisfaisant, mais nous entrons maintenant dans la phase de mise en oeuvre. Dans ce contexte, nos agriculteurs souhaiteraient avoir la certitude

le bilan environnemental de la production ovine est tout à fait convenable. Bref, tous les éléments nous paraissent réunis pour que notre pays joue la carte de l'ambition agricole, en particulier sur le plan de la production ovine.

négociations actuelles de la politique agricole commune, notamment des divers aspects de soutien à la filière de l'élevage, singulièrement celle du secteur ovin.

même si ces filières sont d'ores et déjà en mouvement vers une démarche vertueuse en matière environnementale, il est indispensable de permettre aux producteurs de poursuivre leur culture avec les outils existants, dont fait partie la protection phytosanitaire, en attendant la disponibilité de nouvelles méthodes, telles que les filets dits « » ou la technique d'insectes stériles. Certes, ces filets sont inscrits parmi les aides aux exploitations dans le plan de relance, mais le taux de financement n'encourage pas les producteurs à investir. En ce qui concerne l'introduction de drosophiles stériles, force est de constater que cette technique est prometteuse, mais nous n'en sommes qu'au stade des essais en milieu confiné, bien loin des essais en plein champ. Monsieur le ministre, si cet insecticide venait à être interdit dans les mois à venir, les

au même moment, l'Europe devient importatrice nette de colza et de soja, issus notamment du continent sud-américain, où les pratiques culturales ne sont en rien comparables à celles qui sont autorisées en Europe

en train de travailler ardemment avec la profession sur d'autres intrants qui pourraient être utilisés et qui n'ont pas les mêmes caractéristiques que le phosmet, auquel ils pourraient

vous le savez, un rôle essentiel dans la mise en oeuvre des politiques publiques en faveur de l'égalité entre femmes et hommes, des droits des femmes, de la lutte contre les violences conjugales et de tous les sujets qui nous mobilisent et qui mobilisent la société.

dispositifs. D'autre part, le rattachement au préfet est bien sûr un facteur facilitateur pour les dimensions interministérielles et transversales de la politique publique d'égalité

À ce titre, dans le cadre de la mise en place de la nouvelle organisation territoriale de l'État, les services de ma collègue travaillent actuellement à la revue des missions des équipes territoriales des droits des femmes et à l'égalité, qui ont sensiblement évolué depuis 2017. Je pense notamment aux nouveaux dispositifs issus des mesures prises à l'occasion du Grenelle

L'objectif de cette revue des missions est d'apprécier au mieux les moyens nécessaires à celles-ci et l'organisation la plus appropriée pour les conduire. Cette revue donnera lieu, dans les prochains mois, à une refonte de l'instruction du 3 février 2017,

l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire limite les lieux pouvant accueillir les cérémonies funéraires aux lieux de culte, aux crématoriums et aux cimetières. Les établissements recevant du public qui sont habituellement mis à la disposition des personnes qui souhaitent organiser une cérémonie funéraire laïque sont explicitement exclus des lieux autorisés. ce décret a assoupli les règles, mais uniquement pour lever la limitation du nombre de participants aux cérémonies funéraires dans les lieux de culte. Ainsi, pour les communes, notamment les plus petites, qui ne disposent pas d'un crématorium, cette disposition interdit toute organisation d'une cérémonie laïque dans un lieu clos. Or, en période hivernale, la tenue d'une telle cérémonie en plein air, dans un cimetière- je l'ai personnellement vécu -, peut s'avérer impraticable en raison des intempéries et des températures. lorsque les proches du défunt sont des personnes âgées ou ayant un accès limité à la mobilité, l'existence d'un funérarium à plusieurs dizaines de kilomètres ne représente en aucun cas une solution. Pourtant, les salles mises à disposition par les mairies pourraient tout à fait être soumises aux mêmes contraintes que les lieux de culte. Les maires ont démontré tout leur sens des responsabilités face à la crise sanitaire et ne peuvent être soupçonnés de ne pas pouvoir faire respecter ces consignes dans ce cadre particulier. En outre, aucune donnée scientifique ne vient justifier qu'une salle municipale représenterait davantage de risques, du point de vue de la circulation du virus, qu'un lieu de culte ou un funérarium, d'autant que ces salles sont actuellement fermées à toute autre activité. Avec son projet de loi confortant le respect des principes de la République, visant à lutter contre le séparatisme, le Gouvernement entend proposer des mesures pour contrer ceux dont « l'ambition est de faire prévaloir des normes religieuses sur la loi commune

Aussi, je souhaite demander au Gouvernement de revenir sur le choix réglementaire qu'il a fait, afin que l'ensemble de nos concitoyens, quel que soit leur lieu de sépulture, puissent se voir garantir le droit à une cérémonie funéraire conforme à leurs convictions, y compris en période de crise sanitaire.

touche nombre de personnes confrontées à un deuil. Les membres du Conseil national des opérations funéraires, notamment les représentants des associations familiales, ont souligné combien ce sujet est délicat et combien il a pu être très douloureusement vécu lors de la première vague de l'épidémie de covid-19. Le Gouvernement est attentif à ce sujet ; c'est ce qui l'a d'ailleurs conduit à assouplir, en fin d'année dernière, les conditions dans lesquelles les cérémonies funéraires peuvent avoir lieu pendant la période d'épidémie. Ainsi, en période de confinement ou de couvre-feu, le format des cérémonies funéraires qui demeurent possibles est nécessairement adapté. Ainsi, dans les lieux de culte, une distance minimale doit être assurée : deux emplacements doivent être laissés libres entre deux personnes ou groupes de personnes et une rangée sur deux doit être laissée inoccupée. Dans les crématoriums et les chambres funéraires tout lieu recevant du public ouvert pour la circonstance, il faut également respecter l'obligation d'une place assise libre et d'une distance minimale entre deux personnes ou groupes de personnes. Au regard de sa compétence pour assurer le service public des pompes funèbres et l'équité de traitement entre la crémation et l'inhumation, le maire peut dédier une salle répondant aux exigences fixées pour l'organisation l'organisation des cérémonies funéraires. Toutefois, dans cette hypothèse, compte tenu des dispositions liées à l'état d'urgence sanitaire, que vous avez rappelées, cette salle doit respecter les mêmes contraintes que celles qui sont imposées aux crématoriums. En dehors des établissements recevant du public (ERP), c'est-à-dire dans les cimetières, les cérémonies peuvent accueillir jusqu'à trente personnes. Dans tous les cas, l'état d'urgence sanitaire exige le respect des gestes barrières ; tout moment pendant lequel le port du masque ne peut être assuré de manière continue est évidemment non conforme au respect de ces gestes. Ces conditions restent très douloureuses, nous en sommes

à la dotation politique de la ville (DPV) du chef-lieu du département des Ardennes, Charleville-Mézières, commune de 48 000 habitants. Depuis plusieurs années,

la ville (QPV). Parallèlement à ces actions, des investissements, tels que la vidéoprotection, ont été réalisés pour lutter contre l'insécurité et des projets innovants ont pu être développés, notamment en matière de lecture publique. Au total, entre 2014 et 2020, la ville de Charleville-Mézières a bénéficié, en moyenne, d'une dotation annuelle de 1,3 million d'euros. Néanmoins, en raison de l'introduction de nouveaux critères d'attribution, la ville ne sera plus éligible à la DPV à compter de 2022. En effet, en 2016, la ville n'a pas renouvelé la convention de rénovation urbaine qui lui aurait ouvert de nouveaux droits pour obtenir des dotations au titre du nouveau programme national de rénovation urbaine (NPNRU). Cette décision, prise en accord avec les services de l'État, était motivée par le souci de mener à son terme le programme précédent, conduit entre 2004 et 2018 pour plus de 200 millions d'euros, dont 52 millions d'euros de travaux de voirie et d'équipements, à la charge de la ville. pour avoir voulu achever ses engagements préalables, la ville se trouve lourdement pénalisée, alors qu'il importe de poursuivre la redynamisation des quartiers prioritaires, par des investissements qui portent notamment sur la création ou le renouvellement d'équipements sportifs, pour un total estimé à 21 millions d'euros. Par ailleurs, en complément du soutien aux investissements de la collectivité, la DPV est actuellement mobilisée sur des dépenses de fonctionnement pour des actions innovantes menées dans les trois centres sociaux de Charleville-Mézières. Compte tenu des enjeux démographiques, socioéconomiques et financiers, je me permets de demander que la DPV soit maintenue pour Charleville-Mézières en liaison avec le dispositif spécifique du pacte Ardennes, qui vise à renforcer l'attractivité du département. La

un relâchement de l'effort financier de l'État en faveur de cette commune en particulier, en termes tant de fonctionnement que d'investissement. En matière de fonctionnement,

en enregistrant une augmentation de sa DGF de plus de 750 000 euros depuis 2017. En 2020, son attribution au titre de la DSU a augmenté de 3 %, soit de 400 000 euros, pour atteindre un total de 13,5 millions d'euros. à l'investissement local) déléguée à la région Grand Est en 2020 dépasse 50 millions d'euros. Ce soutien est considérablement renforcé dans le cadre de la relance, avec une majoration de la DSIL qui bénéficiera à la région Grand Est à hauteur de 88 millions d'euros en 2020 et 2021. Monsieur le sénateur, je peux vous assurer que le ministère de la ville est pleinement engagé

Les démarches de soutien mises en place durant la crise se sont également traduites par une enveloppe départementale importante dans le cadre de Quartiers d'été ou encore du fonds Quartiers solidaires, pour un montant de 60 000 euros.

À ce jour, la seule solution connue pour sortir de la crise sanitaire réside dans la possibilité de vacciner le plus grand nombre de personnes. Lors du débat sur la place de la stratégie vaccinale dans le dispositif de lutte contre l'épidémie de la covid-19, le 17 décembre dernier, Bruno Belin insistait sur la nécessité de s'appuyer sur tous les professionnels de santé, notamment les pharmaciens d'officine, qui, à l'exemple des réussites des campagnes vaccinales antigrippales, peuvent proposer et pratiquer la vaccination anti-covid. Deux mois et demi plus tard, nous ne pouvons que nous féliciter du décret publié par le Gouvernement, permettant de répondre à l'urgence de l'accélération de la vaccination. Les pharmaciens sont prêts et habitués aux questions de logistique, de traçabilité et de respect de la chaîne du froid.

tout notre territoire représentent, en ce sens, un maillon essentiel. Les pharmaciens ont déjà prouvé à de multiples reprises leur rôle essentiel ces derniers mois, par exemple pour la distribution de masques, de gel hydroalcoolique ou encore pour pratiquer des tests antigéniques. Depuis le vendredi 5 mars, les pharmaciens d'officine peuvent prescrire prescrire et vacciner les personnes des publics cibles avec les vaccins à ARN messager et à vecteur viral. Le décret pris par le ministre des solidarités et de la santé concerne également les infirmiers, les sages-femmes et les étudiants en santé. En ce qui concerne les pharmaciens, cette ouverture vise d'abord la vaccination en centres de vaccination. À compter de jeudi ou vendredi, l'extension concernera les pharmacies vaccinant contre la grippe et situées dans les 18 départements à la plus forte circulation épidémique, avec une commande, pour cette semaine, correspondant à 67 000 doses. Cette commande est ouverte depuis lundi 8 mars jusqu'à mercredi, Enfin, l'ouverture généralisée de la vaccination à l'ensemble des pharmaciens aura lieu dès la semaine suivante. Comme cela a été indiqué en toute transparence aux représentants des professionnels de santé lors des réunions de concertation, la livraison du vaccin AstraZeneca, qui pourra être utilisé sur le terrain la semaine du 15 mars, est faible : 280 000 doses en tout. En définitive, les pharmaciens auront la possibilité d'injecter 347 000 doses de vaccins au titre des livraisons des semaines du 11 et du 15 mars, à comparer aux 1,6 million de doses pour les médecins. Sous réserve du respect du volume et du calendrier d'approvisionnement par les laboratoires, les commandes seront de nouveau ouvertes à l'ensemble des professionnels de santé susceptibles de vacciner en ville le lundi 15 mars, par une livraison la semaine suivante. Madame la sénatrice, les flux logistiques sur lesquels vous attirez mon attention ne devraient pas connaître de difficultés particulières, étant donné qu'il s'agit d'un réseau déjà éprouvé. Les médecins de ville peuvent, en effet, s'approvisionner auprès des officines de pharmacie et vaccinent depuis le 24 février dernier. De même, les pharmaciens en officine

Madame la ministre, vous n'avez pas répondu à la deuxième partie de ma question, mais je peux comprendre qu'il soit difficile de parler au nom du ministre. J'attire simplement votre attention sur le fait qu'il est important que les pharmaciens hospitaliers puissent vacciner, ce qui constitue une force de frappe supplémentaire. Parmi eux, sont concernés les pharmaciens

et de la santé. Madame la ministre, en mars 2020, alors que notre pays entrait dans la plus importante crise sanitaire de ce siècle, la commune de Loireauxence, en Loire-Atlantique, voyait ses ressources en professionnels de santé s'effondrer. Cette commune nouvelle, qui regroupe plus de 7 700 habitants, a connu, depuis 2018, divers événements qui ont mis à mal son organisation sanitaire et l'accès aux soins de sa population départ à la retraite de deux médecins généralistes et un dentiste, abandon du portage salarial de deux médecins par le centre de santé associatif local et décès brutal d'un médecin généraliste, laissant sans médecin référent près de 2 700 patients. La nouvelle municipalité se saisit pleinement de cette urgence et interpelle les acteurs institutionnels et professionnels, afin de modifier le zonage de médecine générale et d'inscrire la commune en zone d'intervention prioritaire Elle rendrait ainsi son territoire plus attractif au travers des incitations et financements assurés par l'agence régionale de santé (ARS) et l'assurance maladie. À ce jour, au regard des critères retenus par l'ARS et en dépit de la dégradation structurelle et désormais conjoncturelle de l'accès aux soins, la commune semble ne pas être éligible. Pourtant, au vu de la situation, il semble indispensable de réévaluer la situation sanitaire de la commune à l'instant, afin de permettre à ce bassin de population de voir s'installer au moins quatre médecins pour répondre aux besoins.

? La parole est à Mme la ministre déléguée. Madame la sénatrice Meunier, je tiens tout d'abord à souligner qu'en Pays de la Loire, comme c'est la pratique ailleurs, la définition du zonage se fait en concertation avec les acteurs concernés. C'est notamment le rôle du comité technique régional qui valide la méthodologie régionale de définition du zonage. Celle-ci se fait sur la base des données de l'indicateur d'accessibilité potentielle localisée (APL), dont je rappelle qu'il avait été développé pour mesurer l'adéquation spatiale entre l'offre et la demande de soins de premier recours à un échelon géographique fin. Des indicateurs complémentaires régionaux sont également utilisés, comme les installations et départs depuis le dernier zonage. Enfin, le zonage se fait bien évidemment en prenant en compte les retours des comités d'accompagnement territoriaux des soins de premier recours (CATS) sur des réalités de terrain qui ne seraient pas visibles à travers les chiffres : je pense à l'évolution récente de la situation du territoire et à la dynamique de territoire. Pour 2020, en Pays de la Loire, le CTR a validé la proposition de l'ARS de travailler sur des modifications au zonage précédent plutôt que de le redéfinir complètement sur la base des résultats APL 2018. En effet, le risque était était de faire repartir les longues discussions de 2017, qui avaient pourtant permis de trancher certains sujets importants : la maille « bassin de vie » plutôt que l'EPCI, ainsi que l'actualisation des données. Le CTR a donné ses propositions de modification du zonage sur la base des valeurs de l'APL et de leur évolution par rapport à 2018, ainsi que sur les indicateurs complémentaires qui leur ont été fournis. Cela a été fait avec une volonté de soutien aux dynamiques émergentes, en cohérence avec les objectifs du projet régional de santé sur l'accès aux soins. le territoire de Varades, concernant donc la commune de Loireauxence, était classé hors zonage. Il a été décidé de le passer en zone d'action complémentaire (ZAC) du fait de son offre de santé morcelée, plusieurs médecins généralistes avec de grosses patientèles patientèles étant partis à la retraite. C'est donc cette option plutôt qu'un classement en zone d'intervention prioritaire qui a été retenue ; je ne peux vous communiquer tous les arguments qui ont fait pencher la balance dans ce sens et vous invite plutôt à vous rapprocher du CTR. Je souligne simplement que la population ZIP est limitée à 18,2 % de la population régionale, ce qui implique nécessairement de faire des choix. Remettre cette zone en ZIP nécessiterait d'en retirer une autre et de faire un arrêté modificatif, ce qui ne semble pas envisageable dans des délais courts. Je sais néanmoins que les acteurs locaux suivent les évolutions sur le terrain avec une grande attention.

en tout cas, que les élus du territoire seront attentifs à ce type de réponse ; la détermination des élus pourra aussi faire valoir la suite de cette demande. La

Madame la ministre, le 6 octobre 2011, la France a conclu avec le Québec un accord de reconnaissance mutuelle dans le but de faciliter les échanges de masseurs-kinésithérapeutes ainsi que de physiothérapeutes et thérapeutes en réadaptation physique entre nos deux territoires. Cet arrangement a été actualisé en janvier 2014. Cependant, la réforme progressive, en France, du programme de formation en masso-kinésithérapie a rendu cet arrangement inapplicable et, par voie de conséquence, les échanges impossibles. bien sûr dommageable pour les professionnels qui souhaiteraient s'expatrier et, d'une manière générale, pour le dynamisme et l'attractivité de notre système de santé. Cela est surtout problématique pour les jeunes diplômés et pour les étudiants qui se sont inscrits dans des formations en France et au Québec avec l'idée, parfois, de s'expatrier et, souvent, de rentrer auprès des leurs.

Cette situation est évidemment pénalisante pour les personnes concernées, qui attendent, parfois depuis des années, de pouvoir exercer dans leur département d'origine. Elle l'est également pour les territoires ultramarins, dont vous connaissez les faiblesses en matière d'emploi et de démographie médicale. Si des discussions ont cours depuis des années entre les deux ordres et les autorités françaises et québécoises en vue de réviser les termes de cet arrangement et de permettre à nouveau la reconnaissance des qualifications de ces professionnels, aucun accord n'a, à ce jour, été trouvé. Ma question est donc simple : que pouvez-vous nous dire des négociations en cours ? Quand pensez-vous les voir aboutir ? Quelle réponse apportez-vous aux inquiétudes et aux difficultés, parfois matérielles, que rencontrent les jeunes diplômés et les étudiants masseurs-kinésithérapeutes ?

vous le savez, l'arrangement de reconnaissance mutuelle (ARM) concernant les masseurs-kinésithérapeutes, conclu entre la France et le Québec en 2011, établit des procédures destinées à faciliter les échanges de professionnels entre les deux territoires. Il permet aux masseurs-kinésithérapeutes français d'aller plus facilement exercer au Québec et réciproquement pour les physiothérapeutes et les thérapeutes en réadaptation physique québécois. Il prévoit notamment la mise en place de mesures de compensation pour combler les différences substantielles entre ces professionnels, que ce soient en termes de formation ou de champ de pratique. À la suite de la réingénierie du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute en France, organisé en une année d'études communes aux études de santé suivie de quatre ans d'études de masso-kinésithérapie, des discussions se sont tenues entre les autorités québécoises et françaises en vue de réviser les termes de l'arrangement de reconnaissance mutuelle. L'idée était, vous le comprenez bien, d'ajuster les mesures de compensation en fonction des modifications apportées au programme français. Des travaux ont été engagés mais des désaccords entre les parties n'ont pas permis l'actualisation de l'ARM, conduisant à empêcher la bonne application de l'arrangement de reconnaissance mutuelle conclu en 2011. Cette question est donc bien connue et débattue depuis plusieurs années. Le comité bilatéral de l'entente, qui pilote l'arrangement de reconnaissance mutuelle a souhaité, en 2019, constituer un groupe de travail réunissant l'ordre français des masseurs-kinésithérapeutes et l'ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, ainsi que les représentants des ministères français et québécois chargés de la santé. Force est de constater que cette initiative n'a, à ce jour, pas permis aux négociations d'aboutir, malgré l'intervention des ministères et du comité bilatéral de l'entente. Le ministère français des solidarités et de la santé engagera, dans les prochaines des discussions, afin de faciliter la recherche d'un compromis entre les ordres et la négociation d'un avenant à l'ARM existant, qui permettrait aux professionnels de reprendre de reprendre les échanges entre la France et le Québec. À ce stade, il est prématuré de définir les termes éventuels d'un tel accord, mais le ministère veillera au maintien d'un équilibre dans les mesures compensatoires proposées. Il informera bien évidemment la représentation nationale des avancées sur ce sujet.

de l'intérieur. Madame la ministre, dans la nuit du 11 janvier 2021, les pompiers sont appelés à Saintry-sur-Seine pour éteindre un incendie ayant touché quatre véhicules, dont deux appartenant à des agents municipaux. À cette occasion, ils découvrent de très nombreux tags sur les murs de la mairie et ceux de l'école du Parc. Les insultes et menaces de mort taguées visent directement le maire, Patrick Rauscher, nouvellement élu en 2020. En novembre 2020, c'était Aurélie Gros, maire du Coudray-Montceaux, et Baptiste Ollivon, l'un de ses adjoints, qui étaient pris pour cibles avec, là encore, des tags d'insultes sur des panneaux municipaux et des arrêts de bus ainsi que des dégradations de véhicules. Bien d'autres encore, comme, dernièrement, les élus de Corbeil-Essonnes, ont L'autorité est contestée, voir combattue. La démocratie est remise en cause. Le Gouvernement, auquel vous appartenez, madame la ministre, emploie couramment, pour qualifier ces actes, le terme d'« incivilités « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde », disait Albert Camus. Ce malheur pour nous en Essonne, aujourd'hui, c'est l'incroyable message de faiblesse que vous adressez aux fauteurs de troubles. Il est Il est grand temps de prouver à ceux qui commettent ces actes qu'ils seront poursuivis sans relâche et qu'ils seront condamnés comme il se doit. Avec le dernier avatar de Mme la Défenseure des droits, les « zones officielles de non-contrôles d'identité », nous touchons le fond ; une telle déconnexion de la réalité est criminelle. Madame la ministre, à l'instar de ceux de la justice, les effectifs de police et de gendarmerie sont notoirement insuffisants en Essonne pour faire face à la montée de la violence. Qu'envisagez-vous sérieusement de faire, au-delà de simples renforts ponctuels qui ne règlent les choses que jusqu'à ce que les caméras se détournent ?

à la proposition de Mme la Défenseure des droits, qui n'a parlé qu'en son nom propre. Bien évidemment, aucun de nous ne soutient l'idée selon laquelle il y a des endroits dans lesquels il faudrait laisser faire et cesser tout contrôle. Je vous rejoins donc pleinement sur ce sujet.

dit votre opposition à la proposition de Mme la Défenseure des droits. Je vous remercie de saluer les résultats des forces de police et de gendarmerie en Essonne. Je leur rends hommage, elles qui travaillent dans des conditions difficiles. Permettez-moi de vous dire, en responsabilité, sans contester votre action, que notre département est le parent pauvre de la région Île-de-France en termes d'effectifs rapportés à la population. C'est patent

le ministre de l'intérieur. Madame la ministre, ma question concerne la défense extérieure contre l'incendie, souci majeur pour de nombreuses communes de mon département. Le secrétaire d'État Laurent Nunez, que j'avais interrogé en janvier 2020, avait répondu : « J'ai parfaitement conscience que cette réglementation [ ...] peut parfois être contraignante [ parfois] évoluer par le biais de nouveaux échanges avec les partenaires et selon les procédures applicables ». Pourtant, depuis, rien. Un poteau incendie représente 5 000 euros, une bâche, 20 000 euros, une citerne enterrée,

de très petites communes confrontées à ce problème. Sans compter, d'ailleurs, que le débit d'eau n'est pas forcément compatible avec les exigences du schéma. La compétence « eau » revient aux intercommunalités alors que le schéma relève, lui, des communes. Comment faire si le réseau n'est pas modernisé ? Comment implanter les équipements nécessaires sans réserve foncière ? Comment multiplier les sources d'eau dans les communes composées de hameaux isolés ? Tout cela a un coût.

va-t-il rouvrir les échanges évoqués par votre prédécesseur ? Envisage-t-il une évaluation de la mise en oeuvre du référent national dans les différents départements ? Cela me semble indispensable pour prendre en compte les difficultés rencontrées et traiter chaque département à la même enseigne. La parole

sur le terrain, elles peuvent être modifiées, en concertation étroite avec les collectivités territoriales. S'agissant du bilan de mise en place de cette réforme, je peux, d'ores et déjà, vous fournir quelques éléments. Tout d'abord, les premiers règlements départementaux de DECI ont été publiés à partir de 2017. Il convient de laisser le temps nécessaire pour que ce nouveau dispositif puisse produire des effets tangibles. Par ailleurs, les difficultés que vous évoquez ne sont pas communes à tous les départements. Plusieurs services d'incendie et de secours relèvent, en effet, les premières améliorations de la DECI. Nous avons néanmoins parfaitement conscience que cette réglementation, nécessaire pour garantir une lutte efficace et rapide contre les incendies, peut parfois être contraignante dans certaines communes rurales. Comme vous le savez, une mission d'information relative à la défense extérieure contre l'incendie en zone rurale a été créée au sein de la Haute Assemblée. Elle est conduite par les sénateurs Hervé Maurey et Franck Montaugé. La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, chargée de la DECI au niveau national, contribue à ces travaux et réalisera un bilan global de mise en oeuvre

En effet, les périodes de sécheresse et les très fortes chaleurs frappent de plus en plus les zones rurales, comme vous le savez mieux que personne. Elles concernent notamment des secteurs septentrionaux du pays peu habitués à ces situations. Durant ces périodes, les services ont observé une augmentation des feux d'espaces naturels ou agricoles.

Sénat. C'est effectivement un sujet qui nous tient beaucoup à coeur. J'entends que le Gouvernement entend s'appuyer sur ses conclusions, mais nous attendons aussi que vous apportiez vous-même des modifications,

à la suite des dispositions réglementaires qui ont été prises. Les conclusions du dialogue social devaient pourtant apporter une réponse pour tous les personnels du secteur social et médico-social. Ce sont notamment les personnels affectés dans les services de soins infirmiers à domicile (Ssiad), les unités de soins de longue durée (USLD), les établissements et services d'aide par le travail (ÉSAT). Ils sont exclus du Ségur de la santé, contrairement aux personnels relevant de la même filière et du même employeur affectés dans les établissements de santé publics et les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Cette mesure discriminatoire ne semble ni équitable ni compréhensible, au regard en particulier des parcours de vie mis en place aujourd'hui et qui privilégient le maintien à domicile lorsque celui-ci est possible. Ainsi, l'écart de rémunération entre deux agents relevant du même statut, du même grade et du même employeur peut s'élever à 2 100 euros nets par an pour un agent de catégorie C. Cette différence salariale est loin d'être négligeable. négligeable. Il est juste de saluer les avancées du Ségur, mais encore faut-il que celles-ci soient justes. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. De plus, il convient d'ajouter les écarts induits sur les pensions de retraite de ces personnels. Afin de poursuivre le dialogue confiant amorcé au titre du Ségur de la santé, qui doit se prolonger sur les questions de formation de ces personnels, de reconnaissance et d'attractivité de leur profession, de la nécessaire transposition des mesures concernant le public à l'ensemble du domaine médico-social, notamment celui qui relève du secteur associatif, il importe que cette question puisse trouver rapidement une issue favorable. Dans le contexte de crise inédit, où les personnes fragiles et dépendantes sont particulièrement touchées et où tous les personnels affectés à leur prise en charge doivent être reconnus, je vous demande, madame la ministre, quand les dispositions

Mon collègue va dans votre sens : il acte le fait que ce secteur est confronté à d'importantes difficultés de recrutement et de fidélisation des professionnels depuis des années. À l'occasion des accords du Ségur de la santé de juillet dernier, le Gouvernement a institué un complément de traitement indiciaire de 183 euros nets par mois pour les personnels des établissements de santé et des Ehpad, dans un contexte de crise sanitaire, qui, nous le savons tous, a accru les difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs missions. Dans le même temps, le Gouvernement s'est engagé à mener des travaux complémentaires concernant les professionnels du secteur social et médico-social. Ainsi, une mission a été confiée en décembre dernier à Michel Laforcade, ancien directeur Dans ce cadre, la majorité des organisations syndicales, la Fédération hospitalière de France et le Gouvernement sont parvenus à trouver un accord pour revaloriser les professionnels des structures rattachées aux établissements publics de santé, qui, la plupart du temps, partagent les mêmes couloirs que leurs collègues bénéficiaires du CTI. À compter du 1 juin 2021, ces professionnels, qui accompagnent principalement des personnes handicapées ou en perte d'autonomie, bénéficieront de ce nouveau complément de rémunération de 183 euros nets par mois. Celui-ci sera évidemment pris en compte dans le calcul de la retraite. C'est une reconnaissance importante, d'un montant total de plus de 80 millions d'euros pour le budget de l'État, qui sera donc mise en oeuvre chaque année. Par ailleurs, le Gouvernement a demandé à Michel Laforcade d'engager des discussions avec les organisations syndicales s'agissant des professionnels des structures publiques autonomes relevant de la fonction publique hospitalière dès le mois de mars. Je tiens à préciser que, dans le cadre de la mission confiée à Michel Laforcade, sur les métiers de l'autonomie,

Cette mission intégrera l'ensemble des leviers à disposition pour développer la qualité de vie au travail de ces professionnels, améliorer l'adéquation des formations aux besoins des personnes accompagnées et mobiliser l'ensemble des outils des politiques de l'emploi pour favoriser les recrutements. Tels sont, monsieur le sénateur, les éléments que le ministre des solidarités et de la santé souhaitait porter à votre connaissance.

quelques avancées, vous avez bien compris qu'ils ne couvrent pas encore la totalité du champ. J'entends que des négociations sont en cours. Il importe que, face à une même situation professionnelle et un même statut, on puisse obtenir des réponses équivalentes de façon urgente.

un courrier adressé à l'Agence de la biomédecine, sans aucune concertation. Elle est dénoncée par une partie de la communauté médicale, la Coordination de vigilance du groupe hospitalier universitaire (GHU), dans laquelle se retrouvent usagers, syndicalistes, élus de toutes sensibilités politiques, y compris de la majorité présidentielle. Face aux inquiétudes de tous les parlementaires de ce département et à ma demande de rencontre, M. Véran nous a répondu, le 5 mars dernier, en motivant ce transfert par des raisons de sécurité. Utiliser le nombre de transplantations en baisse sans tenir compte de la situation pandémique est plus que fallacieux ! Ce transfert est un vieux serpent de mer, puisque nous avons déjà dû mener une bataille d'ampleur voilà dix ans pour nous y opposer. Nous avions d'ailleurs gagné grâce à la mobilisation des Val-de-Marnaises et des Val-de-Marnais, sous la houlette notamment du président du conseil départemental, Christian Favier, et de la Coordination de vigilance. Madame la ministre, le Gouvernement est-il prêt aujourd'hui à tout mettre en oeuvre pour abandonner ce transfert ?

souhaite porter à votre connaissance le fait que près de 500 patients reçoivent une greffe cardiaque chaque année en France. C'est l'un des domaines d'excellence de nos hôpitaux, dans lequel notre pays ne cesse de se perfectionner et d'innover. Les opérations de greffe cardiaque sont des opérations lourdes, techniques, risquées pour la vie des patients. Elles nécessitent des hospitalisations longues. Au premier semestre 2019, plusieurs opérations de greffe cardiaque réalisées à l'hôpital Henri-Mondor n'ont malheureusement pas permis de sauver la vie de leurs receveurs. Cela a conduit les équipes de cet hôpital et de l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière, qui font tous deux partie de l'AP-HP, à engager une réflexion commune, avec un seul objectif : la meilleure qualité des soins et l'accès de tous aux meilleures pratiques. Cette démarche a abouti à une organisation coordonnée des activités de cardiologie entre les deux sites. Les opérations de greffe cardiaque sont désormais concentrées sur le site de La Pitié-Salpêtrière. Cette organisation doit bénéficier à l'ensemble des patients en attente d'une greffe cardiaque en France, cardiaque en France, tout particulièrement les patients du Val-de-Marne et du sud de l'Île-de-France. Dans cette organisation, le pôle de cardiologie de Mondor est, lui, bien maintenu. Le Gouvernement et le ministre des solidarités et de la santé, par ma voix, en prennent l'engagement. Ce pôle doit poursuivre ses activités en dehors des opérations de greffe, avec une ambition universitaire très forte-

de la communauté médicale. De plus, ce transfert affaiblirait la cardiologie interventionnelle, tout comme l'enseignement et la recherche, et porterait atteinte à l'attractivité générale de cet établissement. Il est très important de prendre cet élément en compte. Au reste, si cette décision était confirmée, elle irait à l'encontre du projet régional de santé

en août dernier, un jeune homme de 25 ans décédait lors d'un stage de survie, dans une forêt du Morbihan, après avoir ingéré une plante toxique, l'oenanthe safranée, cousine de la ciguë. Pourtant, ce stage était supervisé et présenté par son organisateur comme une initiation ouverte à tous les types de publics. suite de ce dramatique événement, l'organisateur a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires. Cette tragique affaire met en fait en lumière le danger causé par le manque de contrôle et d'encadrement de ce type de pratiques, surtout lorsqu'elles sont accessibles aux enfants, Véritable phénomène de société, bénéficiant d'un coup de projecteur avec des émissions de télévision comme, la pratique des stages de survie s'est largement démocratisée au cours de ces dernières années. Ainsi estime-t-on que ce sont entre 100 000 et 150 000 personnes par an qui ont accès à des offres de participation à des camps, stages et séjours dits « survivalistes » en tout genre. Or, actuellement, aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe un cadre juridique spécifique aux stages dits « de survie ». Aucun diplôme n'existe pour attester officiellement des compétences des formateurs qui les encadrent. Certains Certains organismes imposent à leurs instructeurs, pour exercer ces pratiques, une formation équivalente à trois années d'études, avec le Centre d'études et d'enseignement des techniques de survie. Récemment, les principaux acteurs du secteur ont créé le « Cercle de réflexion sur la survivologie

En conséquence, je souhaite, madame la secrétaire d'État, que le Gouvernement soit réactif pour organiser cette réglementation et répondre à la demande de nombreux professionnels. La parole

Selon l'article L. 131-1 du code du sport, les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives. Les fédérations sportives sont constituées sous forme associative, conformément à la loi de 1901. Les statuts restent l'acte fondateur d'une fédération parce qu'ils en définissent évidemment les règles de fonctionnement, mais également les éléments essentiels, comme l'objet, les conditions d'admission ou encore d'adhésion.

Pierre Louault, sénateur d'Indre-et-Loire, n'a pu se joindre à nous ce matin. Il souhaitait interroger le Gouvernement sur la question de la scolarisation en milieu rural, puisque nous sommes au stade de l'élaboration des cartes scolaires pour la prochaine rentrée scolaire. Il est important de tenir compte des difficultés auxquelles sont confrontés les élus dans les zones rurales, notamment lorsqu'ils ont au préalable consenti l'effort de mettre en place des regroupements pédagogiques intercommunaux. Le Gouvernement a fort justement appelé l'attention sur la nécessité de veiller sur la scolarisation des élèves en

dans un contexte de forte baisse démographique, marqué par la perte de 150 000 élèves dans le premier degré. Nous avons dédoublé les classes de CP et de CE1 en éducation prioritaire et nous avons d'ores d'ores et déjà amorcé le dédoublement des classes de grande section de maternelle. En complément, nous avons plafonné les effectifs des classes de grande section, CP et CE1 à 24 sur l'ensemble du territoire. Cela donne la priorité aux savoirs fondamentaux- lire, écrire et compter -, auxquels je sais que le sénateur Louault est extrêmement attaché.

comme dans tous les départements français, le nombre de professeurs pour 100 élèves connaît aussi une nette amélioration, puisqu'il est passé de 5,25 à 5,4 à la rentrée 2020.

Sans action globale, l'épidémie continuera à resurgir partout. Tant que le virus circulera dans une partie du monde, le reste demeurera à risque. La France souhaite augmenter considérablement le budget dédié à l'aide publique au développement. Le débat vient d'avoir lieu à l'Assemblée nationale. Ce n'est donc plus un souhait : c'est une réalité. Nous pourrions alors être en mesure de consacrer assez vite une part significative de ce budget à la distribution de vaccins contre la covid-19 vers les pays en voie de développement. Le Président de la République a d'ailleurs proposé que des mécanismes de partage des doses soient mis en place pour accélérer la distribution des vaccins en Afrique et faire du vaccin un bien public mondial. En effet, l'aide publique au développement permet à l'initiative internationale AMC Covax, portée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), de mettre au moins 1,3 milliard de doses de vaccin à la disposition des populations les plus vulnérables dans les pays Aujourd'hui, alors que la vaccination a commencé dès janvier dans les pays riches, les pays pauvres viennent tout juste de recevoir des doses. Il y a quelques jours, le Ghana est devenu le premier pays, en dehors de l'Inde, à recevoir des doses de vaccin. Cette livraison est la première d'une vague d'expéditions à venir, mais elle a pris du retard. Dans ce contexte, nous avons clairement besoin d'accélérer l'accès aux vaccins. Je souhaite savoir si des fonds supplémentaires sont prévus par la France, parmi les aides allouées à la santé, pour continuer à soutenir le mécanisme international AMC Covax et, le cas échéant, quel sera notre engagement financier dans cette lutte qui doit se faire au niveau international.

La Facilité Covax joue aujourd'hui un rôle absolument essentiel afin d'assurer l'accès équitable aux vaccins partout dans le monde. Plus de 11 millions de doses ont déjà été livrées à travers ce mécanisme, notamment dans

opportuniste une diplomatie vaccinale. La France et ses partenaires européens en particulier sont au coeur de ce projet. Les premiers résultats arrivent. Le Président de la République a lui-même été à l'origine du lancement de l'accélérateur ACT, dont Covax fait pleinement partie. Il a soutenu le multilatéralisme en santé, notamment notamment l'OMS, au coeur de la crise, et appelé à faire du vaccin contre la covid-19 un bien public mondial. La France est, à cet égard, pleinement mobilisée sur plusieurs fronts. Pour répondre plus directement à vos questions, madame la sénatrice, elle contribue aux objectifs de 560 millions d'euros, dont 100 millions d'euros dédiés spécifiquement au mécanisme d'achat de vaccins de la Facilité Covax. Outre les besoins financiers à couvrir pour garantir la pleine efficacité de l'accélérateur ACT, il est absolument essentiel de s'assurer que l'accès équitable et universel universel est bien un objectif central afin de répondre aux besoins mondiaux. Il faut notamment répondre aux différents goulets d'étranglement et faciliter les transferts de technologie pour multiplier les lieux de production, mais aussi obtenir une transparence des prix de la part des industriels. C'est ce que la France a proposé récemment, préconisant, d'ailleurs, dans une charte sur l'accès équitable

les familles, crée une énorme souffrance psychologique et ne peut être que temporaire. Si des mesures dissuasives sont mises en place pour réduire la mobilité, c'est bien l'immunité collective à laquelle nous aspirons qu'il est urgent de mettre en place. À période exceptionnelle, aide exceptionnelle !

tous les acteurs de la culture sont aux abois. Dans ce contexte très anxiogène, certaines structures souffrent plus que d'autres. Dans mon département, l'espace Marcel-Carné, à Saint-Michel-sur-Orge, est dans une situation catastrophique. C'est le maire de cette commune, Sophie Rigault, qui m'a alertée Cet équipement culturel intercommunal, qui compte une salle de spectacle et trois salles de cinéma, est géré par la communauté d'agglomération Coeur d'Essonne Agglomération sous la forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial. Son personnel y est très majoritairement employé sous contrat de droit privé : 15 salariés sur 18 relèvent du droit du travail et la masse salariale représente plus de 40 % de son budget de fonctionnement. Avec la crise sanitaire, cet espace culturel a perdu l'intégralité de ses recettes au guichet, qui constituaient entre 35 % et 40 % de ses ressources. Si le dispositif d'activité partielle a été largement mobilisé par les entreprises de notre pays, il n'a, en revanche, pu être mis en oeuvre par l'espace Marcel-Carné. Peu d'établissements culturels peuvent en effet revendiquer une activité dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources, seuil à partir duquel les salariés peuvent être placés en activité partielle. Je tiens ici à saluer le volontarisme des élus du territoire, qui se battent pour que la culture continue de vivre en Essonne. Je veux aussi souligner l'engagement financier constant des collectivités territoriales, qui ont maintenu leurs dotations budgétaires en dépit des difficultés qu'elles rencontrent. Mais une telle situation n'est pas supportable sur une période aussi longue. Elle est également totalement inéquitable par rapport à celle d'autres structures culturelles ayant opté pour un statut juridique différent, lesquelles ont pu accéder à l'activité partielle grâce à des règles plus souples, alors que les missions de service public exercées sont identiques.

que vous évoquez dans votre question, la France compte de nombreux établissements publics de coopération culturelle qui oeuvrent au quotidien à la démocratisation de la culture sur l'ensemble de nos territoires ; et c'est bien essentiel. Il est vrai qu'ils sont durement frappés frappés par les mesures mises en oeuvre dans le cadre de la lutte contre la pandémie de covid-19. L'ordonnance du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle, modifiée par l'ordonnance du 22 avril 2020, a eu pour objet de limiter les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire des opérateurs publics intervenant dans le secteur marchand. Son champ d'application a été cantonné aux salariés de droit privé des établissements publics à caractère industriel et commercial de l'État et des collectivités territoriales, aux entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l'État, aux groupements d'intérêts public et aux sociétés d'économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire. Je comprends l'importance et l'engagement de Mme le maire Sophie Rigault. s'ajoute une exigence relative à la part de l'activité industrielle et commerciale dans ces structures : elles doivent exercer à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources. Ces conditions complémentaires, vous l'avez souligné, madame la sénatrice, ont eu pour effet d'exclure de nombreux établissements culturels locaux du dispositif de l'activité partielle. Afin de pouvoir accompagner ceux qui sont les plus impactés par cette exclusion, le ministère de la culture a mis en place un fonds de compensation spécifique, d'un montant de 2,15 2,15 millions d'euros, géré par les directions régionales des affaires culturelles. Soyez assurée, madame la sénatrice, de l'entière mobilisation de la ministre de la culture et du regard très particulier de Roselyne Bachelot pour accompagner au mieux ces structures. Elle ne manquera pas, j'en suis sûre, de revenir vers vous, en particulier sur la situation très spécifique de l'espace Marcel-Carné, qui vous tient tant à coeur.

Madame la secrétaire d'État, je souhaiterais attirer votre attention sur la situation des parents séparés ou divorcés dont l'un des enfants est handicapé. L'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les prestations familiales sont dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. En matière d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), c'est donc le principe de l'allocataire unique qui s'applique. En cas de séparation, l'allocation est versée à celui des parents qui bénéficie des allocations familiales ou, si aucun des deux parents n'était allocataire avant la séparation, au premier qui en fait la demande. Les parents d'enfants handicapés qui remplissent les conditions d'ouverture du droit au complément de l'AEEH disposent également d'un droit d'option entre ce complément et la prestation de compensation du handicap (PCH). Pour l'exercice de ce droit d'option, seul le parent allocataire est consulté. Lorsque l'option est choisie, la prestation de compensation du handicap ou le complément de l'AEEH est attribué au seul parent qui bénéficie déjà de l'AEEH. Si la prestation de compensation du handicap peut faire l'objet d'un partage, ce n'est que sur la base d'un compromis entre les deux parents- condition irréalisable en cas de séparation conflictuelle En définitive, l'un des deux parents peut être privé de toute aide, et ce alors même qu'il assume pourtant, de manière alternée, la charge effective de l'enfant. Nié dans sa parentalité, ce parent qui souhaite accueillir son enfant dans un environnement adapté à son handicap devra le financer sur ses deniers personnels. Le handicap ne doit pas être un obstacle à la garde alternée. Le partage des allocations familiales est possible en cas de garde alternée ; les enfants en garde alternée sont bien pris en compte, par exemple, dans le barème de calcul de l'aide personnalisée au logement (APL). Il est urgent d'adapter l'attribution des aides liées au handicap aux situations de garde alternée. Aussi, je souhaiterais savoir ce que le Gouvernement compte faire pour remédier à cette injustice, qui porte préjudice aux enfants en situation de handicap bénéficiant d'une garde alternée.

Babary, les prestations familiales, à l'exception des allocations familiales, ne peuvent aujourd'hui être partagées entre les deux parents dont l'enfant fait l'objet d'une mesure de résidence alternée, en application de la règle de l'unicité de l'allocataire. L'enfant doit en effet être rattaché administrativement à l'un ou à l'autre de ses parents, désigné comme allocataire unique, indépendamment du temps qu'il passe réellement auprès de l'un ou de l'autre. Cependant, les parents ont la possibilité de demander conjointement une alternance de l'allocataire après une période minimale d'un an. Si je partage votre volonté de répartir entre deux parents séparés le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, dès lors qu'ils assument effectivement tous les deux des charges liées au handicap de l'enfant, cette problématique ne concerne pas uniquement l'AEEH et doit faire l'objet d'une étude approfondie dans le cadre d'un projet global de meilleure prise en compte des situations de séparation, pour l'ensemble des prestations familiales. Le partage de l'AEEH est complexe à concevoir et à mettre en place, compte tenu des règles de cette prestation et de ses compléments ; il pose de nombreuses questions de mise en oeuvre. Les compléments de l'AEEH peuvent solvabiliser à la fois une réduction d'activité d'un parent, le recours à une tierce personne ou des frais liés à des soins ou équipements restant à la charge des familles. Cette multiplicité d'utilisations pose des questions complexes de partage de la prestation : une répartition à parts égales serait non conforme à l'équité, puisque c'est souvent un seul parent, majoritairement la mère, qui réduit son activité. Une répartition sur mesure représenterait évidemment une lourdeur accrue en gestion dans l'examen des droits à verser, que ce soit au stade de l'examen initial du droit, mais aussi en cours de versement, notamment si la répartition de la prise en charge des frais change entre les parents. Les questions de partage de l'AEEH pour les parents séparés nécessitent ainsi de réaliser des choix peu évidents, notamment entre simplicité pour l'allocataire, gestion et équité. Ce chantier nécessite donc une analyse approfondie, incluant les autres prestations familiales, afin d'assurer une cohérence d'ensemble des modalités de partage qui seront définies. Un tel partage constituera également un chantier informatique majeur pour les caisses d'allocations familiales et de mutualité sociale agricole. Des travaux sont engagés afin de dégager une solution lisible et équitable entre toutes les familles, quels que soient leur situation matrimoniale ou le mode de résidence choisi pour l'enfant après la séparation, pour la bonne mise en oeuvre d'une telle extension. En ce qui concerne la PCH, le code de l'action sociale et des familles

Les IME sont des établissements essentiels, qui accueillent les enfants en situation de handicap en accueil de jour et de nuit, leur permettant de bénéficier d'un contexte de soins adapté, de scolarité et d'activités permettant un épanouissement personnel. À Lille, que je prends comme exemple parmi de nombreux cas rapportés, l'institut médico-éducatif La Roseraie accueille 105 enfants en semi-internat et en accompagne 20 en

que d'être renvoyés à leur domicile, ce qui les priverait de toute relation avec d'autres jeunes de leur âge, ou d'être accueillis dans des établissements scolaires non adaptés. Comme tous les enfants de la République, ils ont le droit d'être accompagnés, encadrés par des professionnels spécialisés, afin de pouvoir grandir et s'épanouir dans les meilleures conditions possible.

est à Mme la secrétaire d'État. Madame la sénatrice Martine Filleul, vous attirez mon attention sur la réduction du nombre de places dans l'institut médico-éducatif rattaché à l'établissement public départemental de soins d'adaptation et d'éducation. Cet IME est engagé depuis 2019 avec l'agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France dans des réflexions ayant pour objectif d'adapter l'offre aux besoins des territoires. Ces travaux prennent appui sur un état des lieux du public accueilli au sein de l'IME et sur une analyse départementale qui a mis en évidence des besoins importants en matière de prise en charge d'enfants souffrant de troubles complexes. La concertation entre l'établissement, les différents partenaires- éducation nationale, conseil départemental et ARS -a conduit à un projet de transformation guidé par deux grands principes assurer la continuité des accompagnements des enfants accueillis par l'IME et favoriser la diversification de l'offre d'accompagnement. Ces principes s'inscrivent dans le cadre des orientations nationales portant sur la transformation de l'offre et le développement d'une société toujours plus inclusive que porte le Gouvernement depuis 2017. Le projet de transformation de l'IME La Roseraie prévoit ainsi une évolution du fonctionnement de l'établissement en dispositif permettant de déployer l'ensemble des modalités d'accueil modulaire- accompagnement en établissement et par les services en milieu de vie ordinaire. Les accompagnements proposés ont pour objectif d'apporter une réponse graduée et adaptée à la situation de chaque enfant incluant : un accompagnement en service- le Sessad un accompagnement en semi-internat et un accompagnement en internat pour les enfants les plus vulnérables, nécessitant une continuité des soins- il s'agit des 20 places que vous évoquiez. La politique du Gouvernement vise donc à avancer simultanément sur les deux aspects essentiels d'une politique résolument inclusive au bénéfice des enfants et des familles : renforcer l'intervention des professionnels du secteur médico-social au sein des écoles- c'est cette coopération que nous développons -, garantir l'accueil diversifié au sein des établissements chaque fois que nécessaire, et ce de façon plus souple en fonction des besoins. Outre ces évolutions de l'offre,

français. Il existe une convention, signée en 2015 par la France et l'Allemagne, qui stipule que l'impôt sur le revenu doit être uniquement prélevé par le pays de résidence. Or, les frontaliers français placés en chômage partiel par leur employeur allemand en raison de la crise sanitaire subissent depuis lors une double imposition : l'Allemagne, considérant que le chômage partiel est une prestation sociale, applique à ce titre un impôt sur ces salaires. Un accord, conclu le 13 mai 2020 entre la France et l'Allemagne, confirme pourtant que les sommes versées dans le cadre du chômage partiel par les employeurs allemands aux employés français sont imposables dans leur pays de résidence, donc en France. Malgré cet accord, l'Allemagne continue d'appliquer l'imposition de ces revenus, laquelle s'ajoute au prélèvement à la source pratiqué par le système français sur les salaires. Les revenus des frontaliers français sont ainsi doublement pénalisés tout d'abord, par le montant réduit du chômage partiel ; ensuite, par la double imposition qu'ils subissent. Concrètement, un salarié placé en chômage partiel peut perdre jusqu'à 52 % de son salaire Je souhaite donc savoir, monsieur le ministre, comment le Gouvernement peut faire pression sur l'État allemand pour qu'il respecte les accords conclus. Il y a véritablement inégalité devant l'impôt.

je vous confirme que, conformément à la convention fiscale franco-allemande de 1959, modifiée en 2015, les revenus de source allemande versés au titre des indemnités de chômage partiel et perçus par un résident de France ne sont imposables ne sont imposables qu'en France. L'accord du 13 mai 2020 que vous évoquez, conclu dans le cadre de la crise sanitaire liée à la covid, rappelle ce principe. Par ailleurs, comme vous l'indiquez, si ces indemnités ne sont pas imposables en Allemagne en vertu de la loi sur l'impôt sur le revenu, elles sont déterminées selon un mode de calcul prenant en compte la déduction d'un impôt allemand fictif. Une telle déduction a été jugée contraire au principe de libre circulation des travailleurs garanti par le droit de l'Union européenne lorsque, s'agissant d'autres contributions sociales allemandes, la convention fiscale franco-allemande précitée en réservait déjà l'imposition exclusive à la France. C'est pourquoi, pleinement conscient des difficultés que cette situation engendre pour les travailleurs concernés, le ministre Bruno Le Maire a abordé ce sujet avec son homologue allemand, par courrier, l'été dernier. Depuis, nos services continuent d'échanger. Toutefois, le règlement de la situation impliquerait également, et au principal, la coopération du ministère allemand chargé des affaires sociales. Par ailleurs, s'agissant d'une législation prévue par le droit social en Allemagne, plusieurs contentieux individuels ont été engagés par les travailleurs concernés devant les juridictions compétentes de cet État. Je tiens à vous assurer, madame la sénatrice, de la très grande implication de Bruno Le Maire sur cette question, qui doit désormais trouver une solution juste et satisfaisante, sur le plan juridique comme sur le plan économique, et ce dans les plus brefs délais.

Monsieur le ministre, conséquence de la crise économique, le Gouvernement a publié, le 22 juillet dernier, un décret visant à faciliter temporairement la conclusion de marchés publics dans deux secteurs économiques prioritaires : les travaux et la fourniture de denrées alimentaires. Afin de promouvoir la relance, le seuil de dispense de procédures de publicité et de mise en concurrence pour la passation des marchés publics de travaux a été relevé de 40 000 à 70 000 euros hors taxes. Cette mesure est très appréciée des collectivités territoriales, particulièrement des communes et des entreprises qui sont sensibles à la nécessité de pouvoir contracter rapidement des marchés en cette période de ralentissement économique. L'acheteur a ainsi pour seules obligations de choisir une offre pertinente, de faire une bonne utilisation des deniers publics et de ne pas contracter systématiquement avec un même fournisseur lorsqu'il existe plusieurs offres susceptibles de répondre à son besoin. Cette hausse du seuil a été bien reçue par les élus locaux et par les entreprises. En effet, les procédures de passation des marchés publics sont structurellement d'une grande complexité et d'une grande instabilité dans notre pays : montant, objet du marché, circonstances de la conclusion, procédure adaptée ou formalisée Beaucoup d'élus ont du mal à s'y retrouver, d'autant que des normes européennes se superposent aux nationales. La publicité et la mise en concurrence ont de grandes vertus puisqu'elles permettent une égalité de traitement entre toutes les entreprises, une transparence et une saine concurrence pour que l'acheteur public se fournisse au meilleur prix. Mais elles ne sont pas adaptées à toutes les collectivités, particulièrement aux plus petites ou à celles qui n'ont pas forcément des moyens, des services ou des budgets appropriés. Le relèvement du seuil apparaît comme une simplification bienvenue pour de nombreuses collectivités soucieuses de faire travailler au plus vite les entreprises de proximité. Le décret précise que le relèvement du seuil est valable seulement jusqu'au 21 juillet 2021. Afin d'éclairer les collectivités et de donner de la visibilité aux élus, pourriez-vous nous dire, monsieur le ministre, si cette mesure a vocation à perdurer au-delà de cette date ? La

le décret du 22 juillet 2020 portant relèvement temporaire du seuil de dispense de procédure pour les marchés publics de travaux et de fourniture de denrées alimentaires a deux objectifs objectifs : soutenir les entreprises du BTP touchées par les effets économiques de la crise sanitaire en accélérant la conclusion des marchés publics de travaux de faible montant ; lutter contre le gaspillage alimentaire, en facilitant l'écoulement des denrées qui n'ont pu être consommées faute de débouchés. En permettant aux acheteurs publics de conclure des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables jusqu'à 70 000 euros pour les travaux et jusqu'à 100 000 euros pour les denrées alimentaires, ces mesures ont supprimé un formalisme souvent perçu comme excessivement contraignant par les acheteurs de petites collectivités et comme un frein pour les TPE-PME dans leur accès aux marchés publics ; elles ont permis à nos entreprises et producteurs de faire face aux difficultés liées à la crise sanitaire. Toutefois, comme l'a rappelé le Conseil d'État lors de l'élaboration du décret du 22 juillet 2020, parce qu'elles constituent des dérogations aux règles destinées à garantir la liberté d'accès à la commande publique, l'égalité de traitement entre les entreprises et la transparence, ces mesures, justifiées par l'urgence de la situation sanitaire, ne peuvent être que temporaires. Le droit des marchés publics offre aux acheteurs d'autres outils, qui peuvent être mobilisés pour faciliter l'accès de nos TPE-PME à la commande publique et les aider à traverser cette crise, notamment par une définition claire de leurs besoins, la pratique du « sourçage », par un allotissement pertinent ou par l'utilisation de critères privilégiant la qualité ou le développement durable au détriment du critère unique du prix. Afin d'accompagner les acheteurs dans le maniement de ces outils et de sécuriser leur utilisation, le Gouvernement poursuit sa démarche

Par ailleurs, madame la sénatrice, permettez-moi de rappeler que la loi d'accélération et de simplification de l'action publique, dite ASAP, a déjà porté à 100 000 euros le seuil de dispense de procédure pour les marchés publics de travaux jusqu'au 31 décembre 2022. La loi ASAP contient également de nombreuses mesures visant à faciliter l'accès des TPE-PME à la commande publique, notamment dans le cadre de l'exécution des marchés globaux qu'elles ont du mal à remporter.

des comptes publics. Monsieur le ministre, ma question porte sur la compensation de la suppression de la taxe d'habitation pour les syndicats intercommunaux à vocation multiple (Sivom) ayant opté pour la fiscalité additionnelle. Si la loi de finances pour 2020 prévoit le mécanisme de compensation de suppression de la taxe d'habitation pour un certain nombre de collectivités locales, elle ne prévoit pas de compensation spécifique pour les Sivom à fiscalité additionnelle. Dans les Alpes-Maritimes, le Sivom Val de Banquière est particulièrement impacté par cette mesure. Pour la seule commune de La Trinité, par exemple, 400 000 euros ne seront pas compensés dès 2021 ; à Saint-André-de-la-Roche, 130 000 euros

et de la loi de finances pour 2021, j'ai proposé un amendement, largement cosigné par mes collègues du groupe Les Républicains, visant à instaurer une compensation par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement, en prévoyant que son montant évolue en fonction de la valeur locative moyenne des propriétés bâties situées sur le périmètre du syndicat. Lors des débats budgétaires, M. le ministre délégué chargé des comptes publics avait souligné qu'il n'existait pas de problème particulier et qu'il y aurait « un effet de report sur d'autres impositions », notamment sur la taxe foncière et sur la hausse des contributions des communes. Monsieur le ministre, il est impensable pour les maires de devoir, faute de solution trouvée par l'État, augmenter les impôts ou réduire, voire supprimer, les services publics de proximité- je pense à la petite enfance ou aux aides aux seniors -aujourd'hui assurés dans le cadre des compétences déléguées aux Sivom. Où en sont les négociations entre l'administration

le ministre délégué. Madame la sénatrice Estrosi Sassone, comme vous le savez, les syndicats intercommunaux ne disposent d'aucun pouvoir fiscal, ce qui les range dans la catégorie des établissements publics sans fiscalité propre. Le financement du budget d'un tel syndicat comprend une contribution des communes associées, fixée par les communes dans les statuts du syndicat. Lorsque tel n'est pas le cas, le syndicat est compétent pour établir ou modifier la répartition des charges des communes. À titre dérogatoire, le syndicat peut décider de remplacer cette contribution budgétaire des communes par la taxe d'habitation, les taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises. Il s'agit des « contributions fiscalisées Dans ce cas, le syndicat arrête un montant global, réparti dans chacune des communes membres. Cette répartition est proportionnelle aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition.

Non seulement entre-t-il dans le champ de la législation précitée mais, de fait, a-t-il recours à la fiscalisation des contributions. Le recours aux contributions fiscalisées pour son financement résulte donc d'un choix particulier et local d'organisation. Dans la mesure où le Sivom Val de Banquière est assuré de percevoir un montant déterminé de contribution des communes, il n'y a pas matière à compensation dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale. En effet, le syndicat ne perd pas de recettes. La suppression de la taxe d'habitation conduit en revanche à une nouvelle répartition des produits syndicaux entre les contribuables, dont les communes, elles-mêmes compensées du fait de cette suppression, doivent désormais tenir compte dans leurs choix de gestion.

concernant les Sivom. Les maires n'ont pas été élus sur la base d'une augmentation des impôts qu'ils n'ont pas décidée et qui serait imposée d'autorité par l'État ! Véritablement, il est temps de trouver une solution, y compris pour un cas particulier comme celui-ci. La parole est

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord d'avoir une pensée pour mon collègue de l'Oise Olivier Dassault, disparu tragiquement dimanche dernier, alors qu'un hommage lui est rendu en ce moment même à Beauvais. Trumilly, Boubiers, Goincourt, Vandélicourt, Saint-Crépin-Ibouvillers : autant de communes de l'Oise victimes de cyberattaques, avec parfois de lourdes conséquences. Au total, en 2020, selon l'Association pour le développement et l'innovation numérique des collectivités, elles sont plus d'une quinzaine de mon département à avoir été confrontées à ce phénomène inquiétant, qui prend de l'ampleur et révèle des failles importantes de sécurité. Si le contexte sanitaire actuel a accéléré la transition numérique des collectivités et le développement du travail à distance, il a néanmoins eu pour conséquence de rendre plus vulnérables les réseaux des services publics. Pour répondre à cette menace, le Gouvernement va investir un milliard d'euros supplémentaires d'ici à 2025 pour faire monter le niveau général de protection, dans le cadre du plan de relance et du programme d'investissements d'avenir.

quant aux risques numériques. Mais pour les communes de taille modeste, la mise à disposition des outils de sécurisation se heurte à des contraintes financières importantes. La prise de conscience au plus haut sommet de l'État est salutaire. Toutefois, la répartition des moyens de soutien reste floue et la crainte de voir certaines collectivités locales délaissées, comme c'est trop souvent le cas, ne peut, pour l'heure, être complètement écartée. Aussi, monsieur le ministre, quels moyens le Gouvernement entend-il mobiliser afin d'aider, notamment, les plus petites communes à se prémunir contre les cyberattaques ? Envisage-t-il de leur accorder un accompagnement spécifique

Les collectivités territoriales y sont particulièrement vulnérables et présentent la plupart du temps un faible niveau de cybersécurité, dû à une prise de conscience insuffisante des impacts potentiels de cette menace et des bonnes pratiques à mettre en oeuvre pour s'en prémunir. Face à cette menace prépondérante, le Gouvernement a récemment réaffirmé tout son engagement et le Président de la République y a consacré une intervention le 18 février dernier. Il a rappelé la priorité accordée à la cybersécurité de notre pays, en particulier du service public. Concernant le cas spécifique des collectivités territoriales, la réponse est triple. Premièrement, j'évoquerai l'assistance. Il s'agit d'accompagner directement les collectivités dans la résolution d'une cyberattaque et dans la remise en état de marche de leurs systèmes d'information.

Je pense aux prestataires de services qualifiés ou à la plateforme numérique d'assistance aux victimes, cybermalveillance.gouv.fr. Deuxièmement, la réponse est judiciaire. Les récents succès des services d'enquête contre la cybercriminalité organisée, qui ont permis le démantèlement de groupes très actifs avec l'appui de partenaires internationaux, doivent être salués. Ils prouvent l'efficacité de la réponse policière et judiciaire dans le domaine numérique. Si le sentiment d'impunité des cybercriminels est souvent mis en avant, cela ne doit en aucun cas faire hésiter les victimes à porter plainte. C'est en effet indispensable pour mettre fin durablement aux activités de ces groupes cybercriminels. des mesures de prévention. Les services de l'État, en particulier l'Anssi, ont développé un corpus documentaire et technique important pour permettre aux collectivités territoriales de se saisir des questions de cybersécurité et de mettre en oeuvre de nombreuses mesures d'hygiène numérique.